Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, la pratique des fichiers et du fichage est ancienne, mais sa massification et sa banalisation suscitent des interrogations. C'est pourquoi nous avons demandé l'inscription de ce débat à l'ordre du jour du Sénat. Alors que la France a longtemps été un pays où la protection du droit à la vie privée était très forte, on glisse vers une acceptation de la multiplication des fichiers, voire Ainsi, en octobre 2018, le rapport de l'Assemblée nationale sur les fichiers de police dénombre près de 106 fichiers « mis à la disposition des services de sécurité », contre 58 en 2009. Face à ce mouvement effréné de création de fichiers et de récolte de données personnelles, dont la finalité et l'usage réels interrogent, nous avons souhaité l'organisation de ce débat. En effet, nous assistons à une banalisation de l'usage gestionnaire des fichiers par l'ensemble des administrations pour rationaliser les politiques publiques, renforcer la « maîtrise des coûts

l'information générale », et Base élèves, en 2008, ont fait l'objet d'une véritable levée de boucliers. Mais, aujourd'hui, la multiplication des fichiers, dans l'objectif de surveiller, contrôler et réprimer des populations sans réel contrôle parlementaire, se fait dans l'apathie générale. Pire, on accumule ces données dans une logique prédictive, et non préventive. Pourtant, les fichiers sont une maltraitance, un outil de déshumanisation et d'objectivation. Les fichiers ne peuvent pas prendre en compte les singularités, les spécificités de certaines situations. En ce sens, le fichage tend à nier la complexité humaine. Le fichier devient un outil de gestion administrative : on confie à des machines des tâches qui devraient être exécutées par des personnes avec leur conscience, leur savoir-faire, leur capacité d'appréhender des situations particulières. par exemple au fichier Pôle emploi. Créé d'abord pour les demandeurs d'emploi, cet outil sert en réalité à traquer les chômeurs et à accélérer leur radiation. Un service aussi sensible, où l'on connaît les problématiques d'illectronisme ou les difficultés particulières, ne peut être « sous-traité » à un ordinateur. Que dire encore de la création d'un fichier des personnes vaccinées, alors qu'un fichier du nombre de vaccins disponibles et de leur utilisation aurait permis un meilleur contrôle un meilleur contrôle de la politique vaccinale de l'État ? Ainsi, il y a une chosification des gens, mais aussi la volonté de normer les comportements. Il ne s'agit plus de poser des interdits, mais bien d'imposer un comportement, celui que l'État définira comme adéquat. À cet égard, la volonté de ficher les manifestants et les syndicalistes relève moins de la lutte contre les inégalités que de la volonté de discipliner les fractions de la population les plus « indociles Car se savoir fiché ou surveillé empêche l'action, la pensée, et donc l'expression de la démocratie. C'est dans ce cadre que la multiplication des fichiers de police et de surveillance sociale à des fins « sécuritaires » nous interpelle

Ils sont de ce fait susceptibles de violer la présomption d'innocence, le droit au respect de la vie privée et le droit à la protection des données personnelles. Pire, ces fichiers sont souvent faux. Ainsi, par manque d'actualisation ou erreur de saisie, une personne disculpée peut continuer à être enregistrée comme « dangereuse » dans un fichier de police. Les données saisies peuvent peuvent aussi être mal enregistrées, une personne devenant auteur d'une infraction alors qu'elle en est la victime. La liste n'est pas exhaustive ... Ces erreurs peuvent difficilement être corrigées lorsqu'elles se propagent au travers d'interconnexions entre fichiers de police, cette interconnexion complexifiant le droit à la rectification. Or, peu à peu, la sécurité a été érigée en droit en lieu et place de la sûreté. Il ne s'agit plus d'assurer la protection du citoyen, y compris contre l'État, mais de faire de la prédiction de menaces. Nous sommes bien loin du droit à la sûreté, défini par les articles II et VII de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Pas un mois sans qu'une nouvelle idée de fichage sorte des bureaux du ministère de l'intérieur. En février dernier, c'était Gendnote, une application qui facilite la collecte de photos et d'informations sensibles- religion,

qui a pour objet de conserver des informations relatives aux délits routiers et qui, depuis avril dernier, sert de base pour traquer les informations relatives au non-respect du confinement. Que dire encore de l'utilisation illégale des drones et des possibilités de reconnaissance faciale des manifestants ? Or cette multiplication des fichiers de police se fait dans la plus grande opacité et, surtout, brouille la séparation des pouvoirs et la répartition des compétences entre le Parlement et l'exécutif. Le constat fait en 2009 par la mission d'information présidée par Delphine Batho est toujours d'actualité L'exécutif, lorsqu'il entend donner une base juridique aux fichiers de police qu'il crée, peut toujours recourir soit à la voie réglementaire, sur le fondement de l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978, soit à la voie législative. rien n'interdit au Gouvernement de créer un nouveau fichier de police par décret ou arrêté et,, de se soustraire au contrôle du Parlement. Nous pensons que cela doit changer. Ainsi, en 2009, près de 27 % des fichiers n'avaient fait l'objet ni d'une autorisation légale ou réglementaire ni d'une déclaration à la CNIL.

que le Gouvernement a adopté plusieurs décrets pour autoriser l'identification automatique et massive des manifestants, voire la reconnaissance faciale. Cette autorisation s'est passée de tout débat démocratique, comme le souligne La Quadrature du Net. C'est encore par voie réglementaire que, le 2 décembre dernier, trois décrets permettent d'étendre les informations recueillies par les services de police dans trois fichiers qui ont été créés sous la présidence de Nicolas Sarkozy

convictions philosophiques ou religieuses, leur appartenance syndicale, mais aussi certaines de leurs données de santé ainsi que leurs activités sur les réseaux sociaux, le tout pour des finalités élargies qui dépassent la sécurité publique.

Le champ des personnes susceptibles d'être concernées est ainsi très large. Ce faisant, il conduit à stigmatiser la liberté d'opinion, l'action syndicale, le fait d'être adhérent à un syndicat, qui laisserait à penser qu'être adhérent d'un syndicat pourrait être associé d'une manière ou d'une autre à des impératifs de sécurité intérieure, de sûreté de l'État, de lutte contre le terrorisme et les violences urbaines. » En 2011, une personne sur dix était fichée. Qu'en est-il aujourd'hui ? Qu'en sera-t-il demain ? Pire, et c'est une nouveauté, les fichiers pourront aussi concerner des personnes morales ou des « groupements ». On imagine qu'il s'agira d'associations, de groupes Facebook, de squats, de ZAD ou même de manifestations. Enfin, il y a une extension du domaine de la fiche. Jusqu'à présent, les fiches du PASP et du Gipasp ne pouvaient lister l'entourage des « personnes dangereuses » que de façon succincte, sur la fiche principale de ladite personne. Désormais, si la police le juge nécessaire, chaque membre de l'entourage pourra avoir une fiche presque aussi complète que celle des personnes dangereuses, y compris lorsqu'il s'agit d'enfants de moins de 13 ans. En 1983,

d'une autorité grise et pénétrante qui envahit chaque repli de la vie, autorité indolore et invisible et pourtant confusément acceptée. » Pour reprendre ses mots, ne laissons pas l'exigence de sécurité briser le rêve de liberté

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, le sujet de ce débat choisi par nos collègues sénateurs communistes n'est pas dû au hasard, Il trouve sa source dans la parution au, le 4 décembre 2020, de trois décrets modifiant le code de la sécurité intérieure au sujet de trois fichiers de sécurité publique. Naturellement, nous n'ignorons pas que ces décrets ont suscité de fortes inquiétudes de la part de plusieurs associations de défense des libertés, qui redoutent, pour résumer, qu'une nouvelle étape ne soit franchie en matière de surveillance de masse de nos concitoyens. À cet égard, je souhaiterais ce soir que nous tentions collectivement de prendre un peu de recul sur cette question, d'autant que l'essor des fichiers n'est pas un phénomène qu'il serait raisonnable de qualifier de récent. Rappelons-nous du « bertillonnage », qui, au XIX siècle, s'est largement développé afin de rationaliser les techniques policières d'identification, notamment par la constitution de vastes fichiers contenant des données corporelles de nombreuses catégories d'individus : délinquants, criminels, vagabonds, individus soupçonnés d'espionnage ou anarchistes. Il ne nous apparaît dès lors pas incongru que les progrès technologiques changent le visage de ces fichiers de sécurité publique. En premier lieu, ces décrets de décembre dernier procèdent en réalité à une modification du cadre légal afin de prendre en compte l'évolution de pratiques déjà employées par nos différentes forces de sécurité intérieure. Ce nouveau cadre juridique était nécessaire, c'est indiscutable, mais il traduit en creux un besoin opérationnel avéré. S'il fallait le rappeler, ces fichiers ont notamment pour finalité la protection des intérêts fondamentaux de la Nation.

2020, que lesdits fichiers « ne portaient pas une atteinte disproportionnée à la liberté d'opinion, de conscience et de religion, ou à la liberté syndicale en raison de la limitation, par le pouvoir réglementaire, de la collecte et de l'accès aux données concernées « au strict nécessaire pour la prévention des atteintes à la sécurité publique ou à la sûreté de l'État Dès lors, mes chers collègues, je crains que certains d'entre nous ne prennent pour de la peur ce qui n'est rien d'autre qu'une angoisse. Si la peur porte sur un objet déterminé, l'angoisse est une inquiétude vague. L'angoisse est la réalité de la liberté, parce qu'elle en est le possible », écrivait Kierkegaard dans en 1844. Aussi, plutôt que de nourrir une crainte démesurée chez les Français, notre rôle, en tant que parlementaires, est de montrer le chemin vers une plus grande confiance dans nos forces de sécurité et dans leur professionnalisme. L'extension du contenu de ces fichiers ne peut être envisagée comme la porte ouverte à des dérives, qui, si elles se produisent parfois, sont isolées, condamnables et dûment sanctionnées par notre loi pénale. Une telle conception ne rendrait pas justice au dévouement, à la déontologie et à l'éthique de nos fonctionnaires, policiers et gendarmes. La confiance ne nous interdit pas, bien sûr, de nous interroger. Ainsi, concernant le fichier des enquêtes administratives liées à la sécurité publique, qui facilite la réalisation d'enquêtes administratives lors du recrutement d'agents publics à des postes sensibles, le Gouvernement avait répondu à une question écrite de Mme la députée Duriez en 2010 que les données enregistrées dans ce fichier étaient entourées de « garanties renforcées ». Le ministre de l'intérieur expliquait ainsi que « dans les domaines politique, philosophique, religieux ou syndical, ce sont non pas les opinions des personnes, mais leurs seules activités qui peuvent donner lieu à enregistrement, et ce uniquement dans les cas où leur comportement pourrait porter atteinte à la sécurité publique ou s'avérer incompatible avec les fonctions auxquelles elles postulent ». Ce n'est désormais plus le cas. La collecte ainsi autorisée peut se révéler plus attentatoire aux libertés qu'elle ne l'était auparavant. Se pose donc la question suivante : en matière de collecte, les agents candidats un recrutement qui n'ont pas le statut de fonctionnaire bénéficient-ils des mêmes garanties que les titulaires ? Par ailleurs, qu'en est-il exactement de l'interconnexion, autrement dit du rapprochement ou de la mise en relation de ces fichiers avec une ou plusieurs autres bases de données ? En effet, l'interconnexion n'est pas sans incidence en termes d'atteintes à la vie privée, de droit à l'oubli ou encore de présomption d'innocence. Enfin, l'un des enjeux qui doit être au coeur de nos préoccupations est la quête d'une rigueur toujours plus exigeante dans le recueil et la conservation des données engrangées. La fiabilité des fichiers est un gage fondamental de confiance entre l'État et ses administrés. Aussi, quels moyens le Gouvernement met-il en oeuvre pour s'assurer de l'exactitude des informations que l'administration rassemble ? Quels contrôles permettent, le cas échéant, de prévenir ou de corriger des erreurs de saisie, dont les conséquences peuvent être lourdes pour nos concitoyens ? Telles sont, pour les sénatrices et les sénateurs du groupe Les Républicains, les questions qui se posent, madame la ministre, et auxquelles nous vous remercions de bien vouloir répondre.

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, je remercie les élus du groupe communiste républicain citoyen et écologiste d'avoir demandé l'inscription Je souscris totalement à l'intitulé du débat : « Respect des libertés publiques, protection de la vie privée : un nécessaire état des lieux des fichiers dans notre pays. On peut légitimement s'interroger sur les garde-fous et les limites qu'il faut poser pour protéger les libertés fondamentales des citoyens. Pour autant, je ne suis pas certain que nous donnions le même sens à cet intitulé, que nous parlions des mêmes fichiers et que nous visions, en la matière, les mêmes objectifs. Mon collègue l'a rappelé, le 4 décembre dernier, trois décrets ont été publiés afin d'étendre les possibilités policières en matière de fichage.

Pourront être ajoutées des « données de santé révélant une dangerosité particulière, des troubles psychologiques ou psychiatriques », des « comportements et habitudes de vie », des « déplacements », des « pratiques sportives » ou encore des « activités sur les réseaux sociaux Le Conseil d'État, la plus haute juridiction administrative du pays, a rendu un avis positif en amont et il a confirmé sa position quand il a été saisi par des organisations syndicales après la publication des décrets. des décrets. Il s'agit ici de permettre aux gendarmes, aux policiers, aux services secrets, bref à tous ceux qui ont en charge la sécurité des Français,

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, en France, comme dans les autres pays du monde, la lutte contre la crise sanitaire a entraîné une limitation des libertés publiques d'une ampleur inconnue hors période de guerre.

Or ce contexte inédit et exorbitant du droit commun nécessitait précisément qu'une attention vigilante soit portée à l'équilibre subtil des piliers de la démocratie, à la juste proportionnalité entre sécurité des citoyens et garantie des libertés fondamentales, comme préalable à l'exercice républicain. Si votre intention initiale était de protéger la démocratie, les nouveaux contours de l'exercice du pouvoir dessinent un paysage ambivalent, sorte de panoptique géant, où nos libertés sont gravement menacées. Pis, l'emballement des réponses sécuritaires, en muselant les libertés individuelles, nourrit le jeu de ceux qui souhaitent saper les fondements mêmes de la démocratie. Sous couvert de lutter contre le terrorisme, au nom de la sécurité publique, vous avez pris, le 2 décembre dernier, trois décrets élargissant largement les possibilités de fichage et de collecte d'informations. Désormais, tous les acteurs du monde économique, associatif et syndical peuvent figurer dans ces fichiers.

Comble de la surveillance, vous autorisez désormais des pratiques autrefois illégales : pourront désormais figurer dans ces fichiers « les opinions politiques » et les « convictions philosophiques et religieuses » et non plus seulement les « activités » politiques ou religieuses. Une digue importante vient de céder : d'une logique de fichage des activités, on passe à celle d'un recensement des opinions, chacun pouvant être fiché à raison de ses convictions. C'est un acte politique gravissime, pourfendeur de nos libertés fondamentales. Madame la ministre, comment ne pas voir que de tels fichiers légalisent l'intrusion policière dans l'ordre du politique comme dans celui de l'intime, qu'ils entretiennent la confusion entre militantisme, déviance, voire délinquance ?

ceux qui sont susceptibles de porter atteinte à l'ordre public. Toutes ces mesures préfigurent une société gouvernée par la peur, dans laquelle les citoyens seraient privés du droit de penser, de contester, et dont les vies seraient exposées sans limites à la surveillance des forces de l'ordre. La liberté est le droit de faire ce que les lois permettent », écrivait Montesquieu. Considérer que des opinions puissent représenter un danger en elles-mêmes constitue une rupture dans la manière de penser la sûreté de l'État et- ne nous y trompons pas -préfigure l'avènement d'une société de contrôle. Comment, dès lors, ne pas s'opposer à cet arbitraire du fichage, qui fait le terreau du totalitarisme ? Assurer à tous la liberté dans une nation libre, chasser l'arbitraire, faire affirmer et sanctionner cette liberté par une justice libre, telle est l'idée, madame la ministre, que nous nous faisons de la démocratie. Si notre groupe soutient les mesures d'ordre public visant à protéger les citoyens, en accord avec les principes républicains de liberté, d'égalité et de fraternité, il est des principes intangibles trop durement acquis auxquels nous refusons de Dans un pays qui se prétend attaché à la séparation des pouvoirs et à l'État de droit, il est des actes contre lesquels nous devons collectivement nous élever, au nom de nos histoires particulières, de notre histoire à tous, parce que le ferment de notre liberté est celui de notre humanité. Madame la ministre, la protection des citoyens ne peut pas se faire au détriment des libertés publiques. Or vous mettez en oeuvre les moyens de notre futur asservissement, en les offrant à quiconque voudrait demain faire basculer la démocratie. Michel Foucault écrivait en 1975, dans, que le simple fait de se savoir surveillé entraînait une forme d'obéissance.

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, l'article II de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 préfigurait la protection de la vie privée, a ensuite été affirmée en 1948 dans l'article 12 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. En droit français, l'article 9 du code civil, introduit par la loi du 17 juillet 1970, dispose : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée. L'article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne garantit ce même droit. M. le ministre de l'intérieur, Gérald Darmanin, a été auditionné le 12 janvier par la commission des lois au sujet de trois décrets pris le 2 décembre 2020, lesquels avaient suscité une polémique.

utilisé pour contrôler la fiabilité des autorités accédant aux sites sensibles de l'État ; d'autre part, les fichiers de prévention des atteintes à la sécurité publique, pour la police, et de gestion de l'information et prévention des atteintes à la sécurité publique, pour la gendarmerie. conservées les identités d'individus dont l'activité peut porter atteinte à la sûreté de l'État, intéresser l'ordre public ou être en lien avec des faits de violence collective. Contrairement à nombre de fichiers de souveraineté, ces fichiers ont été publiés, ce qui garantit l'information des citoyens et des parlementaires. Ces trois fichiers ont été élaborés entre 2009 et 2011, suivant les recommandations d'experts, puis contrôlés sur leur principe par la Commission nationale de l'informatique et des libertés en 2017 et en 2018. La CNIL définit un fichier comme « un traitement de données qui s'organise dans un ensemble stable et structuré

Ce contrôle a permis de valider ces trois fichiers. Qu'en est-il du contrôle ? Plusieurs associations et syndicats ont demandé au Conseil d'État de suspendre l'exécution de ces décrets modifiant des dispositions du code de la sécurité intérieure. Le Conseil d'État a rejeté l'ensemble des recours, qui portaient sur la conservation et le traitement de données relatives « à des opinions politiques, des convictions philosophiques, religieuses ou à une appartenance syndicale Le Conseil d'État a considéré que « la collecte et l'accès aux données sont limités au strict nécessaire, et ne portent pas une atteinte disproportionnée à la liberté d'opinion, de conscience et de religion ou à la liberté syndicale. Le Conseil d'État, parce qu'il garantit la légalité des décrets, est le protecteur des droits du citoyen et un pilier central de notre République. Nous devons respecter sa décision. De plus, la CNIL vérifie chaque année, en contrôle continu, que les données figurant dans les différents fichiers correspondent bien à la finalité de ces derniers. rappelle également que ces décrets n'ont pas créé ces fichiers, qui existaient déjà. Il s'agissait seulement de préciser les catégories, en tirant les conséquences de délibérations de la CNIL. Resituons enfin leur ampleur : les trois fichiers concernent 60 000 personnes, contre 19 millions pour le fichier de traitement d'antécédents judiciaires, par exemple.

Il est en effet important de ne pas centraliser toutes les données et d'avoir des fichiers distincts et spécifiques, pour chaque type de situation. Cette diversité des fichiers et l'encadrement du recoupement entre eux garantissent le respect des libertés individuelles. Chaque service de sécurité publique a le droit d'accéder à certains fichiers, mais pas à d'autres. Quand ils peuvent accéder à un fichier, c'est seulement pour un objectif précis. En outre, de nombreux fichiers sont constitués par les entreprises privées, notamment les banques, les compagnies d'assurances et, depuis quelques années, les Gafam. Ces fichiers contiennent des informations bien plus détaillées, et souvent plus personnelles, que les fichiers publics. Nous devons donc y être particulièrement attentifs et en assurer le contrôle effectif. Face à ces nouveaux outils, il est bien sûr essentiel d'étendre le domaine du droit et de créer des outils permettant le respect de la vie privée. L'amélioration des démarches de consultation, de rectification et de suppression des données, notamment, grâce à la mise à disposition de lettres types, contribue à cette dynamique. La vice-présidente de la Commission européenne et commissaire européenne à la justice, aux droits fondamentaux et à la citoyenneté, avait posé le 30 novembre 2010 le droit à l'oubli comme l'une des « valeurs » et comme un « droit fondamental » de l'Europe. Toutefois, je veux le redire ici, pour en revenir aux trois fichiers dont je parlais, il s'agit non pas d'étiqueter des personnes selon leurs opinions religieuses, syndicales ou politiques, mais d'identifier les liens entre les individus ayant commis des actions violentes. Disposer de fichiers qualifiés et détaillés est essentiel pour que les outils de renseignement et de sûreté fonctionnent et pour garantir la sécurité publique. Je pense en tout cas,

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, je tiens à remercier nos collègues du groupe CRCE de nous permettre de nous interroger aujourd'hui sur les libertés individuelles et sur la protection de la vie privée de nos concitoyens dans le cadre du fichage. C'est d'autant plus important que la France est plongée dans un état d'urgence- et donc d'exception -quasi permanent depuis la nuit du 13 novembre 2015. Loin de moi l'idée de remettre en cause les raisons pour lesquelles ces lois ont été votées, puis prorogées, tant la folie terroriste qui nous a frappés méritait une réponse forte, mais il est à mon sens nécessaire d'interpeller sur la vigilance, l'exigence dont nous devons faire preuve à l'égard de ces régimes, qui sont, hélas ! devenus la norme. Concernant le régime d'état d'urgence mis en place en 2015, s'il a pris fin en 2017, force est de constater que nombre de ses dispositions sont entrées dans le droit commun. une hausse des prérogatives dévolues au juge administratif, au détriment du juge judiciaire, que ce soit en termes de liberté surveillée ou en cas de fermeture de lieux de culte.

face à de nouvelles formes d'intrusion dans leur vie privée et de fichage. À titre d'exemple, j'évoquerai l'application StopCovid, rebaptisée TousAntiCovid, qui a connu des débuts mitigés et dont l'utilisation se révèle délicate

Je vous épargnerai les remarques sur son incompatibilité avec les systèmes choisis par nos voisins européens. Oui, madame la ministre, la version TousAntiCovid a apporté de la lisibilité et éteint certains doutes.

le temps d'activation moyen du Bluetooth dans la journée, le temps d'ouverture moyen de l'application, le nombre de contacts scorés, le nombre de contacts croisés ». Tout cela sans que l'on sache ni pourquoi, ni comment, ni même dans quel but ... Il y a là de quoi laisser quelque peu perplexe, perplexe, d'autant plus que ce projet de décret supprime également la limite de temps à l'obligation de publication du rapport sur l'application TousAntiCovid. Aujourd'hui, des millions de données circulent chaque jour dans notre pays, des millions d'informations sont collectées nous. Madame la ministre, vous connaissez l'attachement du groupe du RDSE aux libertés, mais aussi son sens des responsabilités lorsqu'il y va de la sécurité de notre pays. Je me permets donc de vous alerter vous alerter sur le fait que toute abdication de liberté, si on veut qu'elle soit consentie, doit être limitée dans le temps. Aussi, nous formons le voeu que, à la sortie de cet état d'urgence sanitaire, nous n'intégrions pas, ou peu, de mesures exceptionnelles dans notre droit commun afin de ne pas fragiliser notre État de droit.

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, à la suite d'Éliane Assassi, j'interviendrai sur les dangers d'un fichage massif des organisations syndicales, des syndicalistes et des militants et d'un fichage politique de l'ensemble de nos concitoyens. Je rappelle la place primordiale des syndicats et du mouvement social dans une démocratie digne de ce nom, au moment où la France est considérée comme une « démocratie défaillante ». Ce rappel est essentiel au moment où il est toujours plus difficile de manifester, d'exprimer des revendications pour plus de justice sociale. Pourtant la mission des syndicalistes est la défense des intérêts individuels et collectifs des salariés. Ils combattent la violence des délocalisations, des fermetures d'entreprises et de plans qui n'ont de sociaux que le nom. Ils dénoncent les privatisations et l'abandon à la finance de biens publics et de fleurons industriels. Ils luttent contre les licenciements indus, pour la préservation des retraites et de notre système de protection sociale, tout en accompagnant des milliers de salariés dans la détresse. Pourtant, plusieurs d'entre eux ont été condamnés à des amendes et des peines de prison à la suite d'actions menées dans le cadre de leurs fonctions syndicales. Ils l'ont été pour s'être opposés à la politique de casse de leur entreprise. Ces condamnations injustes ne suffisent pas au Gouvernement, aujourd'hui le fichage des syndicalistes, au même titre que celui de dangereux délinquants. Il s'agit maintenant de stigmatiser la liberté d'opinion et l'action syndicale. Comment justifier que le simple fait d'être adhérent à un syndicat puisse, d'une manière ou d'une autre, porter atteinte à la sécurité intérieure, à la sûreté de l'État, qu'elle puisse nuire à la lutte contre le terrorisme ou encore, selon les termes des derniers décrets, porter atteinte à l'intégrité du territoire ou aux institutions de la République ? Comment justifier que le droit à résister, à revendiquer, à agir puisse être considéré autre point : la protection des données de santé de nos concitoyens. Aujourd'hui, ces données sont particulièrement convoitées et sont devenues un enjeu majeur. Elles sont par définition particulièrement sensibles, parce qu'elles concernent la santé de la personne, mais aussi parce qu'elles peuvent révéler sa condition sociale ou d'autres particularités personnelles. Pire, ces données pourraient être utilisées à des fins de discrimination : refus d'attribution d'un prêt bancaire, d'accès à un emploi, refus de couverture sociale complémentaire, par exemple en cas de maladie grave. santé, dite Ma Santé 2022, prévoit la création d'une plateforme visant à centraliser l'ensemble des données de santé de millions de personnes, malgré les risques incontestables que présente une telle centralisation. Ces données, qui étaient considérées comme des informations purement médicales dont l'usage était limité aux professionnels de santé ou aux services médico-administratifs, sortent du cadre strict du cabinet du médecin, de l'établissement de santé, pour relever d'un usage plus collectif. En effet, le choix de confier à Microsoft l'hébergement de données permettant de suivre le parcours de santé de 67 millions de personnes sur près de douze années suscite des interrogations, même si le ministre annonçait il y a peu que cet hébergement ne durerait que deux ans,

le Conseil d'État soulignait « qu'il ne peut être totalement exclu que les autorités américaines, dans le cadre de programmes de surveillance et de renseignement, demandent à Microsoft [ ...] l'accès à certaines données outre, l'anonymat du patient n'est pas toujours garanti, ce qui peut encourager des acteurs tiers, tels que des employeurs, des assureurs ou des organismes bancaires, à tenter d'accéder à ces données dans l'objectif de réaliser Comment croire que deux ans ne seront pas suffisants pour que les données, pourtant couvertes par le secret médical, soient bradées ou accaparées par des intérêts commerciaux ou politiques ? Enfin, l'accord national interprofessionnel de 2013 2013 a généralisé les complémentaires santé obligatoires dans les entreprises et ouvert aux assureurs privés l'accès aux fichiers des données de santé des salariés. Les données des réseaux de santé gérés par les complémentaires ne sont pas protégées, ce qui fait peser des risques élevés sur le respect de la vie privée. L'existence des fichiers dans la société a conduit, en 1905, à la démission du gouvernement d'Émile Combes à la suite de l'affaire des fiches, dans lesquelles étaient justement recensées les opinions politiques, syndicales et religieuses des officiers. La généralisation des fichiers dans la société et ses conséquences

madame la ministre, mes chers collègues, jamais en temps de paix nous n'aurons autant porté atteinte à nos libertés publiques les plus essentielles, comme la liberté d'aller et de venir ou la liberté du commerce et de l'industrie. « Pour la bonne cause », me direz-vous, car comme le rappelle le Premier ministre : « Il y a une pandémie qui touche la France. » Dans cette période d'état d'urgence sanitaire, alors que nos préoccupations sont toutes orientées vers la gestion de la crise pandémique et de ses conséquences économiques et sociales, nous devons, mes chers collègues, toujours avoir à coeur de préserver les acquis démocratiques que notre histoire politique et notre doctrine juridique nous ont légués. Selon une étude récente de, les libertés démocratiques ont reflué dans près de 70 % des pays du monde en 2020. Ce chiffre élevé amène à se poser de nombreuses interrogations, surtout quand la France se retrouve dans la catégorie des « démocraties défaillantes C'est pourquoi je rends grâce au groupe CRCE de nous permettre de réfléchir ensemble ce soir à ces questions essentielles et de ne pas nous laisser emporter par le plus grave de tous les risques, celui des accommodements raisonnables, pis, celui de l'accoutumance. Quand le numérique envahit les rapports sociaux à une vitesse incroyable, avec des acteurs privés aussi puissants que des États, se pose toujours avec une grande acuité la question de savoir comment toujours mieux protéger les libertés publiques et la vie privée, quand il faut au même moment lutter contre le terrorisme ou un virus. Légiférons-nous dans le bon sens et avec bon sens lorsque, lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2019, nous avons voté, au Parlement, une disposition donnant la capacité à l'administration fiscale d'aller chaluter des données qui ne sont pas moins personnelles au motif qu'elles sont publiques ? Cette tendance préoccupante, très préoccupante, nous touche nous aussi, législateurs, motivés que nous sommes parfois par le désir d'avoir une administration plus efficace, qui prévient mieux les crimes, les délits et la fraude. Mais que faisons-nous de la vie privée ? Comment préservons-nous ce droit essentiel qui est chahuté dans ses fondements mêmes par les évolutions sociologiques ? Je voudrais vous rappeler ce qu'est la protection de la vie privée, affirmée en 1948 par la Déclaration universelle des droits de l'homme, réaffirmée en droit français à l'article 9 du code civil disposant que : « Chacun a droit au respect de sa vie privée. de sa vie privée. » En 1999, plusieurs décisions du Conseil constitutionnel sont venues étendre cette protection. Évoquer le respect des libertés publiques et de la vie privée, mes chers collègues, nous amène naturellement à nous saisir de la question de l'utilisation des fichiers et de la collecte de données, qui soulève aujourd'hui de multiples interrogations juridiques. Au sens de la loi Informatique et libertés du 6 janvier 1978, ces fichiers constituent des traitements automatisés de données personnelles et font l'objet d'une réglementation spécifique. Même si l'intitulé de notre débat est bien plus large, je concentrerai mon propos sur les fichiers de police et de renseignement. Catégorie à part entière au sein des fichiers administratifs, ils restent spécifiques quant à leur finalité, qui est de participer au maintien de l'ordre public. Cette spécificité les situe ainsi à la frontière entre la répression et la prévention. D'une part, ils sont chargés de collecter des données pour prévenir des atteintes à l'ordre public, quand, d'autre part, ils peuvent être la source de l'action répressive de l'État. Nos concitoyens et, plus largement, les acteurs du débat public dans notre pays n'ont malheureusement commencé à s'intéresser à ces fichiers et à leur finalité, en particulier celle des fameuses « fiches S », qu'à la suite des attentats terroristes survenus depuis 2015. L'utilisation efficace de ces fichiers a souvent permis une réaction rapide dans la recherche des auteurs tout en facilitant l'action répressive, mais a entraîné un débat sur la capacité de l'autorité publique à les utiliser de façon préventive. Ces outils de traitement de données utilisés dans le cadre du maintien de l'ordre ne sont pas sans contrôle. Notre pays dispose aujourd'hui d'un corpus juridique solide qui encadre strictement l'utilisation de ces fichiers depuis une quarantaine d'années. d'y siéger depuis six ans et d'y entamer un deuxième mandat depuis quelques jours, il m'est impossible de ne pas évoquer le rôle crucial de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en la matière. En effet, ces fichiers de police font l'objet d'un contrôle préalable par la CNIL se traduisant par la formulation d'un avis motivé et publié sur l'ensemble des projets de création de ces fichiers. Madame la ministre, à l'occasion du débat de ce soir au Sénat, je me dois aussi d'insister sur le rôle incontournable du Parlement, alors que le pouvoir exécutif continue de disposer de pouvoirs élargis, y compris le pouvoir de légiférer par ordonnance dans de très nombreux domaines. Je ne voudrais pas être inutilement polémique, mais nous allons étudier le mois prochain la proposition de loi relative à la sécurité globale. Ce texte a été écrit sans étude d'impact et sans avis du Conseil d'État. d'État. Il sera l'objet d'une première, puisque, pour la première fois depuis que la loi l'y a autorisé, en 2018, le président de la commission des lois du Sénat a saisi la CNIL d'une demande d'avis sur l'ensemble du texte, et cet avis vient de nous être rendu. Pour la CNIL, le cadre juridique de ce texte, qui contient plusieurs dispositions intéressant directement la protection des données personnelles au travers, en particulier, de la modification du cadre juridique applicable en matière de vidéo et de la réglementation des caméras aéroportées,

Le débat d'aujourd'hui nous donne l'occasion d'évoquer la décision rendue par le Conseil d'État le 4 janvier dernier. Saisie en référé par plusieurs organisations syndicales en raison d'un risque de surveillance de masse, la plus haute juridiction administrative du pays est venue valider trois décrets autorisant les forces de l'ordre à ficher

soupçonnée d'activités terroristes ou susceptible « de porter atteinte à l'intégrité du territoire ou des institutions de la République ». La terminologie retenue reprend d'ailleurs celle du RGPD et de la loi que nous avions débattue et votée ici. Notons que ces décrets avaient en amont fait l'objet d'une consultation de la CNIL, qui avait donné son accord à l'application de ces décrets destinés notamment à lutter contre le terrorisme. Mes chers collègues, force est de constater que, dans la période que nous vivons, sur à peu près tous les sujets, nous observons un recul des libertés publiques, alors qu'elles sont toujours garanties par la Constitution. Plus que jamais, le rôle des magistrats judiciaires et administratifs ou l'existence d'autorités administratives indépendantes comme la CNIL constituent une force, une vigie pour nos libertés.

je tiens d'abord à remercier le groupe CRCE pour ce débat sur le nécessaire état des lieux des fichiers de notre pays. Respect des libertés publiques, protection de la vie privée, voilà les principes qui orientent notre discussion de ce soir. Ce sont des principes largement partagés, à droite comme à gauche, car tout le monde sait que le Sénat est une institution profondément attachée à la défense des libertés publiques. Le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain avait d'ailleurs demandé l'audition du ministre de l'intérieur

Comme citoyens, nous sommes tous fichés de gré ou de force. S'il peut être de bon ton de s'opposer au principe même du fichage, il faut rappeler que nous nous fichons souvent volontairement. Qui, ici, n'a pas adhéré à un Qui, ici, n'a pas adhéré à un parti politique, créé son compte Google, demandé sa carte de sécurité sociale ? Personne, évidemment ! Il faut d'ailleurs reconnaître que nous sommes tous bien moins regardants avec les fichiers détenus par des tiers privés qu'avec les fichiers détenus par l'État. Cela s'explique : rares sont les entreprises à avoir pris le contrôle de pays, créé leur propre police et enfermé des gens selon leurs convictions personnelles., il n'est pas rare que des États dépassent le cadre qu'ils s'étaient fixé il n'est pas rare que des États aient des polices et des prisons à leur disposition. Cela ne signifie pas que l'on doive s'opposer au principe du fichage par les États. Le maintien de l'ordre public, l'accès de tous aux soins, la lutte contre le terrorisme sont des justifications que l'on ne peut nier. Mais c'est ce nécessaire antagonisme entre les besoins de l'État et la défense par les individus des libertés publiques qui fait l'honneur de nos démocraties. Le ministre de l'intérieur doit accepter que les citoyens soient réticents au fichage et les citoyens doivent accepter que l'État satisfasse son besoin d'outils pour la protection de la société. Si je me permets ces rappels, c'est parce que, lors de l'audition de M. Darmanin en janvier, j'avais indiqué, et vous me pardonnerez cette citation : « Ces fichiers semblent de nature à entretenir un climat qui n'est pas sain, en donnant le sentiment de contrevenir aux libertés publiques. » M. Darmanin m'avait répondu, courroucé : « Je ne peux pas laisser dire que les décrets contreviennent aux libertés publiques. » Au-delà de la joute oratoire, je tiens à dire au Gouvernement qu'il a l'obligation de laisser dire aux parlementaires tout ce qu'ils veulent. Très bien ! Pour ma part, j'ai été étonné, dans sa réponse d'alors, par l'interprétation que le ministre a faite de l'avis de la CNIL. Ainsi, M. Darmanin a déclaré devant la commission des lois : « [Les fichiers] ont été validés par le Conseil d'État et la CNIL en amont, et de nouveau par le Conseil d'État en aval. Ils sont d'autant plus respectueux des libertés publiques qu'ils ont été conçus à la demande de la CNIL. » Il se trouve que la commission des lois a aussi auditionné la présidente de la CNIL, Mme Marie-Laure Denis, la semaine dernière. Cette dernière a déclaré- cela figure au compte rendu de la commission des lois - Une évolution sémantique a eu lieu : on est passé d'activités politiques, religieuses, philosophiques et syndicales, à des " opinions politiques ", des " convictions philosophiques et religieuses " et " l'appartenance syndicale

celui-ci vise à éclairer le pouvoir réglementaire ou le législateur et il appartient au juge administratif de se prononcer sur la légalité des actes réglementaires. En l'espèce, le Conseil d'État s'est prononcé en référé, sans déceler de doutes sérieux sur la légalité du texte, mais il aura très certainement à se prononcer au fond. En tout cas, au fond. En tout cas, le collège de la CNIL ne s'est pas prononcé sur l'évolution sémantique. » Exactement ! Le Gouvernement souhaite-t-il répondre à cette déclaration de la présidente de la CNIL

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, la conciliation entre le droit de l'individu et le droit de la société, entre l'ordre public et la liberté, n'est pas un problème récent. En droit français, l'article 9 du code civil dispose : « Chacun a droit au respect de sa vie privée. » À l'origine de cette demande de débat, on retrouve les trois décrets du 2 décembre 2020 et la tribune publiée le 17 décembre dernier dans le quotidien : « Extension des fichiers de renseignement : un nouveau danger pour nos libertés. Cette tribune, signée par de nombreux élus de gauche et écologistes, dénonçait l'atteinte à la démocratie et le mépris du Parlement. S'il s'agissait bien d'une compétence réglementaire et non législative, l'élaboration de ces décrets aurait toutefois pu donner lieu à une consultation du Parlement, ou à tout le moins à une communication. Au lieu de cela, les parlementaires en ont appris l'existence par voie de presse, après leur publication. Une telle manière de procéder est incompréhensible. Elle l'est d'autant plus lorsque l'on se souvient des débats suscités par le décret Edvige en juin 2008. Ce décret créait un fichier recensant les personnes « ayant sollicité, exercé ou exerçant un mandat politique, syndical ou économique ou qui jouent un rôle institutionnel, économique, social ou religieux significatif ». Il fut finalement retiré au mois de novembre suivant. Ce manque de transparence nourrit malheureusement les suspicions envers l'État de droit. Aujourd'hui, via les réseaux sociaux, tout le monde est fiché par des Big Brother privés, sans rien y trouver à redire. Le constat est sans appel : pour les Français, il est aujourd'hui plus facile de s'inscrire sur Facebook ou Instagram que de télécharger l'application TousAntiCovid.

Si le fichage étatique effraye, c'est en raison des conséquences que l'État pourrait en tirer, mais le fichage est parfois nécessaire et certains fichiers ne seront jamais contestés. On peut citer pour exemple le fichier des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes, ou encore celui sur les agréments des assistantes maternelles, dont la création vient d'être annoncée. La sécurité ne figure pas au nombre des libertés, mais elle est bien l'une des conditions de leur exercice. Pourquoi ces récents décrets alarment-ils ? Parce qu'ils s'inscrivent dans une logique de prévention des risques. Il s'agit d'un fichage d'opinions, de convictions et non de comportements répréhensibles. Ces décrets prévoient en effet la création de fichiers de police pouvant contenir des données relatives « à des opinions politiques, des convictions philosophiques, religieuses ou une appartenance syndicale », ainsi que des données « de santé révélant une Le premier est le fichier EASP, pour « enquêtes administratives liées à la sécurité publique », utilisé avant le recrutement de fonctionnaires sur des postes sensibles. Il s'agit d'éviter de recruter des personnes potentiellement dangereuses ou radicalisées. Les deux autres fichiers sont le PASP, pour « prévention des atteintes à la sécurité publique », et le Gipasp, gestion de l'information et prévention des atteintes à la sécurité publique ». L'un, le PASP, est géré par la police, l'autre, le Gipasp, par les gendarmes.

Soumis pour avis à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, ils font l'objet de recours contentieux. Le 4 janvier dernier, le Conseil d'État a jugé qu'il n'y avait pas lieu de prononcer leur suspension. Selon le juge des référés, la collecte de ces données dans les traitements litigieux n'entraîne pas d'atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie privée ou à la liberté d'opinion. Deux arguments ont retenu son attention. D'une part, seules les activités « susceptibles de porter atteinte à la sécurité publique ou à la sûreté de l'État pourront donner lieu à l'enregistrement de données. D'autre part, il sera interdit de sélectionner dans le traitement une catégorie particulière de personnes à partir des seules données sensibles. Jusqu'au jugement au fond de ces affaires, ces fichiers sont donc légaux. Mais tout ce qui est légal est-il souhaitable ? La question que l'on peut légitimement se poser est la suivante : en quoi le fait de ficher des opinions, y compris philosophiques, peut-il garantir la bonne tenue d'une manifestation ? Élargir le fichage, c'est considérer que des opinions puissent représenter un danger en elles-mêmes. Cela représente une rupture importante et inquiétante dans la manière de penser la sûreté de l'État. En 2009, Robert Badinter déplorait déjà le recours presque obsessionnel à des fichiers, et s'interrogeait sur cette dérive inquiétante consistant à passer « d'une justice de liberté à une justice de sûreté ». Un tel changement de doctrine ne peut être accepté que si l'on peut s'assurer de son utilisation et de son effectivité. Pourra-t-on s'assurer que les personnes fichées seront pleinement informées et pourront exercer leur droit de rectification ? Quelles conséquences légales seront tirées de ces fichiers ? Pourront-ils justifier une arrestation ou un non-recrutement ? La parole

Madame la présidente, madame la ministre, chers collègues, la pandémie mondiale de la covid-19 a vu émerger la prolifération de virus d'un autre type : les virus informatiques. Les établissements de santé, les laboratoires de diagnostic ou de recherche sont régulièrement victimes de piratages. Les données de santé sont très prisées ; récupérées, elles sont revendues à prix d'or. À titre d'exemple, la société Moderna a été touchée par une cyberattaque en juillet dernier AstraZeneca en a été victime en novembre. Plus récemment, en janvier, l'Agence européenne du médicament confirme qu'une version falsifiée des fichiers volés chez Pfizer a bien été partagée sur le. La CNIL La CNIL a publié en janvier un avis sur plusieurs mesures mises en place par le Gouvernement dans le cadre de la crise sanitaire. Cet avis a mis en évidence plusieurs manquements dans la gestion des données personnelles, notamment sur leur durée de conservation et leur sécurité dans le logiciel de. Pour la Pour la CNIL, bien que prévu par une circulaire, ce processus de entraîne une dispersion des données dans les messageries. De plus, ces informations, en partie stockées sur des serveurs, sont conservées trop longtemps, faisant fi du règlement général sur la protection des données personnelles.

elle estimait que l'application ne pouvait être déployée que si son utilité pour la gestion de la crise était suffisamment avérée et si certaines garanties étaient apportées. Son utilisation devait être temporaire et les données devaient être conservées pendant une durée limitée. Insidieusement, TousAntiCovid tend vers les mêmes travers, sans vigilance particulière sur la durée et sur les conditions de stockage des informations personnelles. Les appels à la vigilance sont nombreux. En janvier 2021, Christian Babusiaux, l'ancien président de l'Institut des données de santé, appelait le Gouvernement à rompre au plus vite le contrat conclu avec Microsoft pour la construction d'un grand entrepôt d'hébergement des données de santé. Les doutes sur les garanties offertes par le droit américain font craindre pour la sécurité des données de santé des Français, avec un risque d'exploitation abusive de ces dernières. Si le Gouvernement s'est engagé à retirer l'hébergement de ces données à Microsoft d'ici à deux ans, ce délai est trop long au regard des risques d'exploitation des données à d'autres fins que celles pour lesquelles elles ont été communiquées. Enfin, en décembre, le Gouvernement avait présenté un projet de loi instituant un régime pérenne de gestion des urgences sanitaires. L'article 1 de ce texte prévoyait de subordonner le déplacement des personnes et l'exercice de certaines activités à la présentation d'un test de dépistage ou au suivi d'un traitement préventif, y compris la vaccination- en d'autres termes, la mise en place d'un passeport sanitaire. Si le projet de loi a depuis été retiré et son examen renvoyé après la sortie de la crise, une telle mesure doit être envisagée avec la plus grande prudence. Nous veillerons au respect des libertés individuelles, le Parlement est garant de cette protection, en s'appuyant sur les avis de la CNIL. Dans son avis, la CNIL rappelle ainsi que les données de santé sont protégées par le secret médical et ne doivent être traitées que par des personnes habilitées et soumises au secret professionnel. Vous l'aurez compris, madame la ministre, la protection des données personnelles est un enjeu majeur, les données personnelles de santé ; elles doivent être strictement protégées pour garantir la liberté de chacun. Ces données statistiques destinées à une exploitation collective pour la recherche ou l'industrie sont particulièrement convoitées et font l'objet d'espionnage industriel ou de sabotage malveillant. Il est de votre responsabilité et de celle du Gouvernement de les protéger efficacement, de veiller à ce que leur utilisation ne soit pas dévoyée, de garantir notre indépendance nationale en la matière.

de fichiers dans notre pays, en particulier ceux liés à l'utilisation des données de santé, qui tendent à se généraliser : je pense notamment au dossier médical partagé. La

Mesdames, messieurs les sénateurs, je me réjouis de la tenue de ce débat et de pouvoir participer à vos échanges très riches sur ce sujet fondamental du respect des libertés publiques, de la protection de la vie privée et du nécessaire état des lieux des fichiers dans notre pays.

Premièrement, un contexte sécuritaire qui s'est globalement tendu, avec une menace terroriste désormais structurante. Deuxièmement, des évolutions techniques et technologiques qui ouvrent de nouvelles potentialités de traitement des données. Troisièmement, un droit des données qui n'a cessé de s'étoffer et de se préciser, avec notamment l'entrée en vigueur dans notre droit du règlement général sur la protection des données de 2018, sa transcription dans la loi Informatique et libertés que vous connaissez bien. C'est de ce triple mouvement qu'est issue la situation que nous connaissons aujourd'hui. Elle se caractérise, me semble-t-il, par de nouveaux besoins des services de sécurité en termes d'accès aux fichiers, d'interconnexion, de fiabilisation des identités des personnes inscrites, d'exigence accrue de transparence et de précision, cela a été mentionné à plusieurs reprises, sur chacun sur chacun des fichiers, sur leurs finalités, leurs modalités de fonctionnement, les mesures prises pour s'assurer que ne sont collectées et conservées que les seules données strictement nécessaires. J'observe une J'observe une forme d'exigence contradictoire à l'égard de l'État, cela a été dit également. Les Français, et c'est heureux, sont de plus en plus sensibilisés aux enjeux de leurs données et du traitement qui peut en être fait. Ils sont aussi parfois méfiants envers des fichiers mis en oeuvre par l'État et singulièrement par le ministère de l'intérieur. Dans le même temps, il me semble que les Français attendent aussi des policiers et des gendarmes qu'ils puissent anticiper, prévenir les menaces, agir, détecter dès que possible les individus potentiellement dangereux, travail quotidien pour lequel le recours aux fichiers est bien souvent, chacun le comprend, indispensable. À cet égard, la demande croissante d'enquêtes administratives sur des personnes exerçant des métiers sensibles de la sécurité, mais aussi de l'enseignement, de la santé et des services publics est révélatrice. Dans ce contexte, nous avons fait le choix, en France, de conserver un régime de fichiers de sécurité très protecteur. En effet, alors que le RGPD et la directive Police-Justice de 2018 régissant les fichiers dont nous débattons ce soir ont inauguré un vrai changement de paradigme, notamment en supprimant le régime de déclaration d'autorisation des fichiers, nous avons fait le choix de maintenir un régime d'autorisation pour les fichiers de sécurité. Cela signifie que tout traitement de données à caractère personnel qui intéresse la sûreté de l'État, la défense ou la sécurité publique, ou qui a pour objet la prévention, la recherche, la constatation et la poursuite des infractions pénales, l'exécution des condamnations et des mesures de sûreté, doit être autorisé par un acte réglementaire pris

après avis de la CNIL. D'ailleurs, les décrets qui ont été évoqués apportent des actualisations sémantiques sur ces questions, je tiens à le préciser. Chacun des fichiers du ministère de l'intérieur doit donc respecter les dispositions cardinales du droit des données personnelles. Ces données doivent être collectées et traitées de manière loyale et licite- c'est le principe de légalité ; elles doivent être collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes- c'est le principe de finalité ; le responsable d'un traitement ne peut enregistrer ou utiliser des informations sur des personnes physiques que dans un but précis, légal et légitime elles doivent être adéquates, pertinentes, non excessives au regard des finalités recherchées- c'est le principe de proportionnalité et de pertinence. Les informations enregistrées doivent donc être strictement nécessaires au regard de la finalité donnée et connue du fichier. Elles doivent être exactes, évidemment, et tenues à jour. Toutes les mesures raisonnables doivent être prises pour que les données à caractère personnel inexactes, eu égard aux finalités pour lesquelles elles sont traitées, puissent être effacées ou rectifiées, et ce sans tarder.

Concrètement, chaque fois que le ministère de l'intérieur envisage de créer ou, le plus souvent, de modifier un traitement de données à caractère personnel, il doit d'abord prouver à la CNIL,

Pour ce faire, le ministère doit notamment réaliser une analyse d'impact relative à la protection des données dans laquelle il expose très précisément ce qu'il veut faire et quelles dispositions à la fois juridiques et organisationnelles il prendra pour assurer que

au regard des exigences qui pèsent sur chaque responsable de traitement ; contrôle externe par la CNIL, qui mène aussi régulièrement des contrôles sur les traitements de données de la police et de contrôle du juge, en l'occurrence le Conseil d'État, saisi de nombreux recours contentieux. Dans ce contexte juridique en pleine mutation, les auteurs du rapport d'information de la commission des lois de l'Assemblée nationale consacré aux fichiers de sécurité intérieure, en 2018, saluaient 2018, saluaient la diffusion, au sein de la police, comme de la gendarmerie, d'une véritable culture des libertés individuelles. Notre enjeu, aujourd'hui et demain, est bien là : respecter pleinement un droit exigeant, un droit protecteur des données et des libertés publiques, tout en donnant aux services les moyens en leur permettant d'être pertinents et réactifs. Je voudrais préciser que nous parlons là de 65 000 personnes, c'est-à-dire bien moins que le rapport de un sur onze évoqué

a demandé au Gouvernement, dont ce n'était pas l'objectif initial, de procéder à une évolution terminologique pour mieux tenir compte de la rédaction actuelle de la loi Informatique et libertés qui désigne les données sensibles. J'espère ainsi apporter une réponse aux interrogations du sénateur Jérôme Durain. Durain. Jusqu'à présent, il était précisé, par exception à l'interdiction de collecter des données sensibles, qu'il était possible de réunir dans ces fichiers des données concernant les « activités » politiques, religieuses, syndicales. La traduction française du RGPD ayant retenu, pour qualifier les données sensibles, les termes « opinions », « convictions » et « appartenance », le Conseil d'État a tout simplement souhaité s'aligner sur cette rédaction. Ces éléments peuvent être importants pour contextualiser la menace. Savoir qu'un individu adhère, par exemple, à des thèses antispécistes est important pour contextualiser des faits de dégradation de commerces ou de sites de production alimentaires auxquels il incite à participer. Il s'agit d'une contextualisation. De même, le militantisme n'est évidemment pas, en soi, une donnée intéressant les services au regard d'un engagement syndical. En revanche, il est important de savoir si un individu radicalisé est représentant du personnel de l'entreprise : dans ce cas, il peut jouir d'une influence plus forte auprès de ses collègues pour les inciter, par exemple, à rejoindre des idéologies prônant la violence, voire à passer à l'acte. L'examen du Conseil d'État intervenant après l'examen de la CNIL, il me semble normal que celle-ci ne se soit pas prononcée sur cette évolution. Les décrets précisent explicitement qu'aucune recherche dans les fichiers ne peut être réalisée à partir de ces données sensibles. de ces données sensibles. Le Gouvernement ne permet pas le fichage des syndicalistes. Appartenir à un syndicat n'est jamais une raison justifiant un fichage.

être fichés, et c'est heureux. Un membre du Conseil d'État, chargé de la vérification, remet chaque année un rapport sur ce sujet. J'espère avoir ainsi répondu à l'interpellation de Mme la sénatrice Assassi. Il n'y a pas non plus d'interconnexion automatique entre les différents fichiers.

tous les jours à Google ou à différents acteurs numériques sont bien plus sensibles, bien plus personnels et bien moins contrôlés. Je voudrais enfin préciser que des personnes morales peuvent, à l'évidence, représenter une menace

Dans ce cas, le fichage se fait au travers des individus qui les composent. Elles ne figureront donc pas comme élément d'évaluation de la menace que représente une personne. Toutefois, le fait qu'un individu participe, par exemple, aux réunions d'un groupe néonazi constitue en soi une information, un élément d'appréciation de sa potentielle dangerosité. De même, il peut être important de signaler qu'une personne présentant une menace fait partie d'une association ou d'un groupement quelconque pour déterminer, par exemple, son potentiel cercle d'influence, ses relations, ses tentatives d'entrisme ou de déstabilisation. En matière de lutte contre le terrorisme islamiste, il est absolument fondamental de pouvoir disposer de ces informations, très précieuses pour les forces de sécurité intérieure.